Très bien ! Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, d'habilitation à prendre par ordonnances

plus-value s'élève à 1,129 million d'euros. Elle a été réalisée grâce à une flambée boursière en faveur de Danone faisant suite à l'annonce de la suppression de 900 emplois. Ce point est extrêmement grave sur le plan éthique et, peut-être, sur le plan juridique : de par vos fonctions, vous avez organisé ce plan social et vous en avez récolté les fruits pour votre profit personnel. De là à parler d'initié, il n'y a qu'un pas à franchir

du code du travail, dont la conséquence sera la précarisation et l'appauvrissement de milliers et de milliers de salariés. Le plafonnement des indemnités de licenciement en est un exemple concret. Madame la ministre,

Ce qui est ciblé ici, c'est le travail de nuit, et le Gouvernement saisit une nouvelle fois l'occasion de déréguler un peu plus le code du travail. Comme chacun le sait, le travail de nuit est aujourd'hui réglementé et limité par la loi aux cas exceptionnels : continuité du service public, obligation de maintien de la production, Il présente des contreparties obligatoires en matière de repos et de rémunération. La période de travail de nuit correspond aux horaires effectués entre 21 heures et 7 heures du matin. Le recours au travail de nuit suppose la conclusion d'un accord collectif, et je rappelle que les règles qui l'encadrent ont été considérablement modifiées, successivement par la loi Macron et par la loi El Khomri.

que de mesures assez techniques. Mais pourquoi n'avoir pas envisagé d'élargir ce qui définit actuellement la période de nuit plutôt que de la restreindre ? Cela ne constituerait-il pas une vraie valeur ajoutée pour les salariés ? Comme vous le savez, dans notre pays, environ 3,5 millions de personnes travaillent de nuit, soit 15,4 % des salariés. Personne ne peut nier l'impact de ces horaires atypiques sur la santé : troubles du sommeil, augmentation du risque du cancer du sein, etc.

sont de nouvelles protections des salariés qui sont laminées. Vous comprendrez que nous demandions, au travers de cet amendement, la suppression de cet alinéa 22. Une vraie mesure sociale aurait été de proposer la limitation du travail de nuit. Ce n'est pas le choix que vous avez fait : dans ce domaine, vous ouvrez encore un peu plus la brèche de la déréglementation,

Des effets avérés sur le sommeil, des effets probables sur la santé psychique, des performances cognitives diminuées, l'obésité, le diabète, les maladies coronariennes, le risque de développer un cancer : voilà, mes chers collègues, la liste des conséquences avérées du travail de nuit sur la santé des salariés. Si l'Organisation mondiale de la santé, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, le Conseil économique, social et environnemental, le Centre international de recherche sur le cancer s'accordent pour donner l'alerte sur les risques qu'entraîne le travail de nuit, alors il est de la responsabilité du législateur d'en limiter les cas de recours. À ces risques sanitaires s'ajoutent des conséquences sociales pour les travailleurs concernés, qui vivent à un rythme décalé de la majorité de nos concitoyennes et concitoyens. Demandez à une infirmière qui travaille la nuit comment elle concilie son métier avec sa vie familiale et sociale ; pourtant, elle est bien obligée de Pour toutes ces raisons, nous nous opposons fermement à ce que le travail de nuit soit facilité, en particulier s'il s'agit, comme nous le craignons, de répondre à une demande de commerces ouverts tard le soir. Nous estimons que le travail de nuit doit rester exceptionnel et limité à certains secteurs d'activité. C'est pourquoi nous demandons la suppression de l'alinéa 22.

Tourenne. Le travail de nuit est gravement nuisible pour la santé, chacun le sait. Il est démontré depuis longtemps que la durée de vie des personnes qui ont travaillé de nuit est réduite, ainsi que la durée de vie en bonne santé. permettez-moi de citer deux sources. En 2007, le Centre international de recherche sur le cancer a ajouté le travail posté à la liste des agents probablement cancérogènes. De son côté, dans son rapport du 22 juin 2016, l'ANSES affirme que les risques de troubles du sommeil et de troubles métaboliques sont avérés. Il existe des risques probables de cancer, d'obésité, de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires, de troubles psychiques, et cette liste n'est sans doute pas complète ! La proposition de soumettre le caractère exceptionnel du travail de nuit à la négociation collective est donc particulièrement inquiétante. Le travail de nuit n'est déjà que trop répandu. Il a malheureusement en partie perdu son caractère exceptionnel. Mais ce caractère exceptionnel est un élément de la protection sanitaire du monde du travail. À ce titre, il est un principe d'ordre public sanctionné par l'article L. 3122-1 du code du travail.

Nous connaissons tous l'arrêt, grande enseigne des Champs-Élysées, en vertu duquel « le travail de nuit ne peut pas être le mode d'organisation normal du travail au sein d'une entreprise et ne doit être mis en oeuvre que lorsqu'il est indispensable à son fonctionnement ». le Gouvernement entend revenir sur cette jurisprudence en « créant une forme de présomption de légalité du recours au travail de nuit dès lors que l'entreprise peut s'appuyer sur un accord collectif autorisant cet aménagement du temps de travail ». voté, contre notre avis d'ailleurs, une présomption de légalité de l'accord collectif. En d'autres termes, il suffirait qu'un accord soit obtenu dans une entreprise, conclu par des délégués du personnel non mandatés ou par référendum sur l'initiative de l'employeur pour que le travail de nuit soit présumé légal. Il est aisé d'imaginer en quels termes la question serait en réalité présentée aux salariés et les conditions dans lesquelles un accord favorable au travail de nuit serait obtenu. On voit, dans ces conditions, ce qu'il adviendra d'un principe d'ordre public protecteur de la santé des salariés. Pour ces raisons, nous sommes opposés à l'introduction de cette disposition dans la loi. Très bien ! L'amendement n° 66 rectifié,

Le travail de nuit peut avoir un caractère exceptionnel. Il doit effectivement être encadré en fonction des professions et en priorité par les accords de branche. Toutefois, si le travail de nuit n'est pas « naturel c'est le terme qu'il faut employer -, eu égard au rythme biologique de l'être humain, il n'a pas nécessairement de caractère exceptionnel. Il est inhérent à certaines fonctions, comme la continuité du service public, la sécurité et un certain nombre d'autres activités.

notamment pour assouplir à la marge la plage horaire du travail de nuit. Nous pourrons ensuite modifier, si nécessaire, l'ordonnance lors de l'examen du projet de ratification.

L'article L. 3122-1 du code du travail, tel que modifié par l'article 8 de la loi Travail, pose comme principe d'ordre public que le travail de nuit est exceptionnel. Son recours doit prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, et il doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale, ces deux notions n'étant pas définies par la loi. loi. En même temps, l'article L. 3122-15 du code du travail renvoie à un accord d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, à une convention ou à un accord collectif de branche, le soin de justifier le recours au travail de nuit. Le cadre juridique actuel n'est donc pas satisfaisant, ce qui explique sans doute le manque de cohérence de la jurisprudence, qui a dû combler les lacunes de la loi.

il convient de distinguer l'activité d'une entreprise, qui peut être normalement et habituellement effectuée la nuit, du travail des salariés la nuit, qui doit rester exceptionnel dans son principe. La loi n'interdit pas le travail de nuit, mais elle l'encadre pour éviter sa banalisation. Cet équilibre a paru justifié à la commission des affaires sociales.

Cela étant, le Gouvernement souhaite sécuriser les entreprises qui ont recours au travail de nuit tout en veillant à protéger la santé et la sécurité des salariés dans un cas de figure précis. Tout d'abord, la plage horaire du travail de nuit couvre la période comprise entre 21 heures

Le départ effectif des salariés a donc lieu après 21 heures, sans pour autant que l'employeur ni d'ailleurs les salariés perçoivent cette situation comme relevant intégralement du régime du travail de nuit.

De plus, le Gouvernement souhaite sécuriser le recours au travail de nuit. À cette fin, il entend le présumer justifié, notamment au regard de son caractère exceptionnel, en le faisant reposer sur l'accord des partenaires sociaux. conforme à la celle qu'a prise la cour d'appel de Nîmes dans un arrêt rendu le 22 septembre 2016 à l'occasion d'un recours contre un accord d'établissement qui a adopté une interprétation laissant davantage de place à la négociation collective et à la présomption de justification sous réserve de cette négociation collective. Il faut donc faire confiance aux partenaires sociaux, qui connaissent mieux que quiconque la nécessité de recourir ou non au travail de nuit, qui- j'insiste sur ce point -conservera son caractère exceptionnel.

Il ne s'agit en rien d'augmenter considérablement le nombre de salariés concernés. Il s'agit simplement de sécuriser à la marge les entreprises lorsqu'elles recourent au travail de nuit. Pour ces raisons, je suis défavorable aux amendements n 127, 157 et 46 rectifié.

comment faire en sorte que, de manière ponctuelle, les compétences de certains salariés soient utilisées dans d'autres entreprises afin d'en assurer le fonctionnement pour telle ou telle problématique ? Comme chacun le sait, le prêt de main-d'oeuvre est une procédure autorisée, mais assez précisément définie par le code du travail. ailleurs, il est évident que l'entreprise utilisatrice doit, dans un premier temps, s'être tournée vers d'autres modes de recrutement de personnels extérieurs, notamment au réseau des agences d'intérim. Que signifie donc « favoriser et sécuriser », pour reprendre les termes de cet alinéa ? S'agit-il, comme nous sommes tentés de le croire, de favoriser le nomadisme professionnel plus ou moins organisé par les directions d'entreprise et de groupe en revenant, autant que faire se peut, sur l'abondante jurisprudence qui a souvent établi son caractère illicite ? S'il s'agit de cela, pourquoi offrir cette nouvelle « souplesse »

partager le souhait des auteurs de l'amendement d'assouplir les règles encadrant le recours au temps partiel, que nous dénonçons d'ailleurs ici depuis plusieurs années, mais cet amendement tend un nouveau sujet à la liste déjà longue des points sur lesquels le Gouvernement nous demande de l'habiliter à prendre des mesures par ordonnances. Son adoption constituerait, selon la commission, un élargissement du champ de l'habilitation et serait ainsi contraire à l'article 38 de la Constitution.

dans les entreprises de moins de cinquante salariés, sans pour autant diminuer les garanties et les protections offertes aux salariés concernés. Cette disposition, qui figurait dans l'avant-projet de la loi exonère les entreprises de l'obligation de conclure un accord collectif pour mettre en place cette forme d'organisation du travail. Toutefois, ces entreprises devront se soumettre aux conditions introduites par la loi Travail pour assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés en forfait, c'est-à-dire un suivi renforcé de l'activité et un contrôle, sous la responsabilité de l'entreprise, de l'adéquation de la charge de travail avec les temps de repos. Une telle mesure est particulièrement intéressante pour les entreprises innovantes en phase de croissance,

le précédent, contraire à l'article 38 de la Constitution. L'une des pistes pour encourager le développement des conventions de forfait est l'élargissement des accords de branche, qui lui est prévu à l'article 4 du projet de loi.

même lorsqu'elles ne sont pas en mesure, comme les TPE et PME, de négocier et de conclure un accord collectif sur ce point.

récente fait état d'une chute libre du nombre d'affaires soumises à la justice prud'homale. Quelles en sont les causes ? Est-ce le signe qu'un plus faible nombre de cas prêtent à contentieux ? Non

la suppression des juridictions de proximité. Elles ont ainsi augmenté les embouteillages dans le traitement des affaires. Pour raccourcir les délais d'instruction, il n'est pas nécessaire de limiter l'accès au juge : il faut simplement renforcer leurs moyens. Vous obtiendrez alors une justice efficace et de proximité. Pierre Joxe s'est exprimé récemment

qu'il ne suffit pas de modifier le régime fiscal et social des sommes versées en cas d'indemnités abusives ; il convient également de simplifier le régime applicable, devenu beaucoup trop compliqué. En effet, si l'on souhaite encourager la conciliation, il faut créer des règles fiscales et sociales simples et attrayantes, ce qu'elles ne sont pas toujours aujourd'hui. Les règles qui se sont superposées

Il est en effet préférable de résoudre les conflits qui peuvent survenir entre un employeur et son salarié par la voie de la conciliation, plutôt que d'en arriver à la voie juridictionnelle. Elle est donc défavorable

heureusement, ils sont aidés par les syndicats -, on fait en sorte que ce soit de plus en plus en plus difficile ! Madame la ministre, j'ai bien compris que vous n'étiez pas favorable

Toutefois, face à l'inertie et la rigidité des outils conçus au fil du temps, il est utile, même urgent, de revoir la politique d'insertion dans l'emploi des personnes handicapées pour éviter l'augmentation des inégalités et les trappes à exclusion que représentent trop souvent l'inaptitude au la qualité de travailleur handicapé, la RQTH, et la désinsertion professionnelle. Pour ce faire, il faudrait que, grâce au dialogue social renforcé, les politiques publiques soient réellement décloisonnées,

et que toutes les parties prenantes concernées soient sollicitées systématiquement et suffisamment tôt. En effet, les pouvoirs publics doivent veiller à la participation des personnes handicapées, ainsi que des représentants et des proches de celles-ci, au processus de décision. Enfin, une stratégie pluriannuelle devrait être définie, intégrant l'objectif de réduction du chômage des travailleurs handicapés et d'accès de ceux-ci à un emploi de qualité, avec le déploiement de données et de règles de connaissance à partager dans la transparence. C'est à ces conditions que les parcours vers et dans l'emploi seront sécurisés pour tous. Le Président de la République a fait du handicap l'une de ses priorités. Cette priorité ne peut être à la marge, à l'opportunité d'un volet handicap ou d'une communication bienveillante. Elle doit s'inscrire dans la continuité et dans la mise en oeuvre des grandes lois d'affirmation des droits imprescriptibles des personnes handicapées, dans le cadre d'une politique inclusive unissant toutes les politiques publiques.

plan de santé au travail, approuvé par l'ensemble des partenaires sociaux, prévoit des actions spécifiques pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Devant le COCT, le Conseil d'orientation des conditions de travail,

pour objet d'offrir aux primoarrivants une première prise en charge à visée médicale, la prévention de l'introduction sur le territoire national de pathologies infectieuses en provenance de pays tiers relevant davantage du contrôle sanitaire aux frontières. Il est donc proposé de remplacer l'expression « contrôle médical », qui qualifie de manière inadéquate cette activité de l'OFII, par l'expression, neutre, de « visite médicale », mieux à même d'accompagner l'évolution de cette mission.

... Certains secteurs très concurrentiels, notamment du nettoyage, ont mis en place avec les partenaires sociaux des modalités pour préserver l'emploi en organisant le transfert des personnels

le domaine de la propreté. Je rappelle que certaines conventions collectives contiennent des stipulations obligeant l'entreprise qui remporte un nouveau contrat avec un client à reprendre l'ensemble des salariés de l'entreprise évincée, dès lors qu'ils travaillaient sur le site du client. La Cour de cassation a toutefois considéré, le 15 janvier 2014, que les transferts conventionnels ne constituaient pas une raison objective et pertinente justifiant une différence de rémunération entre salariés.

Cette disposition exclut donc du bénéfice de l'indemnité de licenciement, quel que soit le niveau de celle-ci, une partie non négligeable des salariés, alors même qu'un licenciement marque toujours une rupture dans la vie professionnelle du salarié, qu'il intervienne au bout de quelques mois ou de plusieurs années. elle induit des effets de seuil très importants pour les salariés licenciés disposant d'un peu moins d'une année d'ancienneté. Le présent amendement a pour objet de permettre au Gouvernement d'abaisser, voire de supprimer, la condition d'un an d'ancienneté nécessaire à l'ouverture de droits à l'indemnité de licenciement, étant

Sur le fond, l'amendement vise à permettre au Gouvernement de faire bénéficier de l'indemnité légale de licenciement des salariés ayant moins d'un an d'ancienneté. Il offre donc potentiellement de nouveaux droits aux salariés.

mais en demandant à Mme la ministre de veiller à ne pas alourdir excessivement les charges pesant sur les entreprises, surtout les petites, en augmentant de manière inappropriée le montant de l'indemnité légale par voie réglementaire.

est à Mme Laurence Cohen. Actuellement, les entreprises ne sont pas dans l'obligation de présenter un plan de sauvegarde de l'emploi lors de licenciements économiques effectués à la suite d'un refus de modification du contrat de travail quand le nombre d'emplois concernés est inférieur à dix dans la durée d'un mois.

dix salariés » par les mots « plusieurs salariés ». Ainsi, il deviendra beaucoup plus difficile de déguiser un licenciement économique de plus de dix salariés en le fractionnant en plusieurs licenciements de différents types et en l'étalant sur la durée.

La loi prévoit que les règles du licenciement collectif s'appliquent au-delà de dix-huit licenciements économiques sur une année civile et au-delà de dix licenciements sur une période de trois mois consécutifs.

refusant la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail est calqué sur le seuil des licenciements collectifs, dont le régime est prévu aux articles L. 1233-21 et suivants

par le juge dès lors que l'information et la consultation ne revêtent pas un caractère loyal et sincère ou lorsqu'elles ne comprennent pas un effet utile lié à la consultation. Vous l'avez compris, cet amendement s'inscrit dans la suite logique de l'amendement que j'ai défendu ici même hier, et qui visait à interdire les licenciements présentés comme économiques, alors qu'ils sont en réalité uniquement motivés par des intérêts particuliers, les intérêts exclusifs des actionnaires. Tandis que certains se gavent de stock-options, de dividendes à la hausse,

de la loi relative à la sécurisation de l'emploi en 2013. Le législateur avait alors fait le pari de confier aux syndicats et aux employeurs le soin de fixer

Cet amendement créerait plus de difficultés qu'il n'en réglerait. M. le rapporteur a rappelé la réforme menée en 2013 : le fait

Enfin, vous évoquez, mais trop vaguement, le périmètre à prendre en considération pour apprécier les moyens du PSE, alors qu'il est clairement défini. En effet, le PSE est apprécié au regard des moyens dont disposent les entreprises. Si l'entreprise appartient à un groupe, le PSE est apprécié au regard des moyens du groupe, tel qu'il est défini à l'article L.

en leur permettant d'élaborer des propositions complémentaires ou alternatives aux projets de l'employeur. Nous suggérons également que ces propositions soient sérieusement considérées, mises à l'étude et en débat par l'employeur. Cela permettrait aux représentants du personnel et de se constituer en pouvoir de contre-proposition effectif, au besoin. Il s'agirait là d'une évolution indéniable dans la prise en compte des salariés, et d'une évolution positive pour toutes les parties prenantes. En parallèle, nous proposons un renforcement des pouvoirs du comité d'entreprise en cas de recours par l'entreprise à des formes précaires de contrat de travail. L'avis conforme du comité d'entreprise serait requis, afin de prévenir de manière efficace le développement de contrats atypiques au sein du collectif de travail,

l'amendement de notre collègue Christian Favier, il pourrait à l'avenir formuler des propositions complémentaires ou alternatives au projet de l'employeur. Ce serait une évolution majeure de notre droit, dont nous ne mesurons pas toutes les conséquences, et qui doit être conciliée avec le pouvoir de direction de l'employeur.

a force de loi et s'applique à l'ensemble des salariés du secteur, y compris celles et ceux dont les entreprises ne sont pas adhérentes aux branches. Il s'agit d'une procédure importante pour les salariés des TPE et PME qui n'ont pas de représentants syndicaux, comme cela peut être le cas, en particulier, pour les employés du secteur des services à domicile, dont on connaît les conditions précaires et flexibles de travail. Depuis la loi relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale de 2014, une ou plusieurs organisations patronales, dont les entreprises adhérentes emploient plus de 50 % des salariés des entreprises affiliées, peuvent déjà s'opposer à un accord de branche. Ouvrir la possibilité de s'opposer encore

voulez prendre en compte les objectifs de la politique économique et sociale. Mais, dans les faits, ce sont principalement les accords de branche sur les salaires qui ont permis aux salaires de continuer à augmenter en France malgré la crise. Et vous voulez les faire voler en éclats ! Ce n'est pas en créant de nouveaux droits pour les salariés que vous porterez atteinte à la compétitivité des entreprises françaises. Bien au contraire, cela permettrait d'améliorer leur rentabilité, même si vous le réfutez malheureusement

Primas, sur l'article. Je vais évidemment émettre une opinion assez différente. L'article 4 aborde la question de l'extension et de l'élargissement des accords. Aussi me semble-t-il utile, au nom de ma collègue Élisabeth Lamure, de rappeler les conclusions de l'étude que la délégation aux entreprises a fait réaliser l'an dernier par l'institut allemand IFO pour comparer les pouvoirs et la représentativité des représentants de salariés dans l'entreprise en France et en Allemagne. Cette étude montre notamment les incidences économiques de l'organisation du dialogue social. L'IFO indique qu'en France, l'extension quasi automatique des accords collectifs par l'État et par le ministre du travail, donc, aboutit à un taux de couverture de la négociation collective de 98 %, soit un chiffre bien plus élevé que le taux de salariés travaillant dans des entreprises membres d'une organisation patronale. patronale. En Allemagne, ces deux taux sont équivalents et s'établissent autour de 57 %. Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, ce taux de couverture des conventions collectives est seulement de 23 %, la procédure de l'extension y étant plutôt rare. L'IFO est très critique à l'égard de l'extension à la française, tant en termes d'effets sur le chômage, puisqu'elle renforce la dualité du marché du travail, que d'effets sur la concurrence. D'ailleurs, je rappelle que le Conseil d'État a déjà censuré l'extension de stipulations portant une atteinte excessive au principe de la libre concurrence. Analysant les propositions du rapport Combrexelle, l'IFO a même suggéré de supprimer l'extension des accords de branche par le ministre du travail, afin de stimuler la concurrence et d'encourager la création d'emplois. Les petites entreprises nous le confirment : elles ont besoin de plus de marges de manoeuvre. Elles souhaitent notamment pouvoir conclure des accords d'entreprise, même en l'absence des délégués syndicaux : c'est la deuxième priorité mise en avant par les chefs d'entreprise que nous avons rencontrés sur le terrain,

alinéas ne me semblent pas poser de problème majeur. Le quatrième alinéa tire les conséquences des nouvelles dispositions en matière de représentation patronale à la suite de la loi de 2008 et du regroupement d'organisations dans l'U2P, alinéa se situe dans la même perspective quant au fonctionnement et au financement du fonds paritaire. Il appartient aux organisations représentatives de régler ces questions. alinéa traite de l'élargissement d'un accord collectif, procédure qui permet au ministre du travail de rendre obligatoires, dans un secteur géographique ou professionnel qui n'a pas conclu un accord de branche depuis au moins cinq ans, les stipulations d'une convention de branche déjà étendue dans un secteur analogue. Cette disposition est en rapport avec le regroupement et la réorganisation des branches qui sont en cours. Elle est intéressante pour les petites entreprises qui pourront ainsi être couvertes par un accord. En revanche, l'alinéa 2 vise à améliorer et sécuriser juridiquement l'extension des accords collectifs en précisant les conditions dans lesquelles les organisations représentatives d'employeurs peuvent s'y opposer et en réaffirmant les pouvoirs du ministre, ce qui concrètement pose question. C'est la loi du 5 mars 2014 qui, en fixant les règles de représentativité des organisations patronales, a créé un mécanisme d'opposition à l'extension d'un accord de branche sur leur initiative. madame la ministre, pouvez-vous nous indiquer ce que vous entendez exactement par « améliorer et sécuriser juridiquement le dispositif d'extension », ainsi que vos pouvoirs en la matière ?

l'objet de cet article 4 ? Il organise tout simplement la suppression du principe d'extension, c'est-à-dire la possibilité d'étendre le bénéfice d'un accord collectif à l'ensemble d'une branche professionnelle. C'est pourtant

donc pas de course à l'abaissement des conditions de travail dans ce secteur d'activité. C'est cet acquis du Front populaire qui a contribué à l'uniformisation actuelle des conditions sociales des travailleurs d'une même branche. ailleurs, et en totale contradiction avec ce que j'évoquais précédemment, l'article prévoit la possibilité d'une extension extra-branche. En résumé, une entreprise ne serait plus obligée d'appliquer l'accord de sa branche et pourrait appliquer l'accord d'une autre

En effet, il est de mon avis qu'une telle mesure contraindra et musellera le dialogue social au sein des entreprises. L'adoption de ces réformes en procédure accélérée et par ordonnances ne me semble pas judicieuse si l'on souhaite réellement renforcer le dialogue social. Alors que la majorité des effets de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ne sont pas encore évalués, il paraît peu opportun de modifier les règles qui exonéreraient certaines entreprises d'accords collectifs ou de conventions collectives.

à l'intérieur de notre territoire. Nos économies ont déjà suffisamment souffert et continuent suffisamment de souffrir de la concurrence déloyale en partie causée par les exigences de la mondialisation

d'État autorise et même impose dans certains cas au ministère de prendre en compte une atteinte excessive à la concurrence et à l'intérêt des tierces parties à l'accord. Par exemple, dans le secteur de l'assainissement et de l'eau, un arrêté d'extension a été annulé sur ce motif. Il s'agit ici de faire respecter les règles de la concurrence entre

Monsieur le président,

Le périmètre de la branche peut être utile, mais uniquement à la condition que les entreprises adhèrent pleinement aux conventions qui y sont négociées. Le seul périmètre à prendre en compte doit être celui des entreprises. C'est à cet échelon que tout se joue.

Le scrutin est ouvert.

En effet, pour quatre des dix critères, c'est un retour en arrière, avec une vision médicalisée et restrictive de la pénibilité, bref le contraire d'une politique de prévention pour des personnes qui manipulent des charges lourdes, subissent des postures pénibles, des vibrations mécaniques, ou sont exposées à des risques chimiques. On nous dit que c'est l'expertise médicale qui décidera si elles doivent rester à leur poste. Or obtenir la reconnaissance taux d'incapacité de 10 % s'assimile souvent à un parcours du combattant. Quant aux autres, elles partiront en bonne santé à la retraite- du moins le croient-elles -, mais elles seront rattrapées quelque temps plus tard par le déclenchement d'une maladie. Donc, pas de prévention et pas davantage de réparation : c'est la double peine pour certains travailleurs qui ont le nombre d'années d'incapacité le plus élevé et l'espérance de vie la plus courte. Revenir sur ces critères, c'est aller à l'encontre d'un principe de justice et de lutte contre les inégalités. Car, rappelons-le, les inégalités de santé se constituent principalement dans le monde professionnel. Vous proposez même de modifier l'intitulé de la réforme en effaçant le mot « pénibilité », ce qui pourrait signifier : « Cachez donc ces conditions de travail que nous ne saurions voir ! Il semblerait que certains considèrent que l'emploi du mot « pénibilité » induit que le travail serait une souffrance. Bien sûr qu'il l'est, pour des centaines de milliers de Français,

est-ce un signe de bien-être au travail ou est-ce un signe de pénibilité ? S'il vous plaît, nommons les choses telles qu'elles sont, sans occulter de tristes réalités ! Le psychanalyste Jacques Lacan avait raison d'écrire que ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Nommons ces choses-là, car elles existent, et n'en ayons pas honte

Vous envisagez de supprimer quatre des dix critères prévus : la manutention des charges lourdes, l'exposition à des postures pénibles, à des vibrations mécaniques ou à des risques chimiques. Pis, vous changez le principe même du dispositif initial pour les six critères restants. Vous préférez guérir plutôt que prévenir

donc de rattraper un déséquilibre face à la vie, souvent lié au milieu social dont est issu le salarié. Pourquoi un ouvrier qui vit en moyenne moins longtemps qu'un dirigeant de grande entreprise ne pourrait-il pas partir plus tôt à la retraite, d'autant qu'il ne qu'il ne bénéficiera ni du même montant de ressources ni du même état de santé pour en profiter ? Je ne veux pas, mes chers collègues, faire ici l'apologie de la lutte des classes. Néanmoins, les études sur les inégalités à la naissance et les chiffres sont têtus. Par ailleurs, vous changez radicalement le mode

cesser de faire contribuer les cotisations patronales au financement ? Ne subsiste, dans votre projet de réforme, ni le fond ni la forme du compte pénibilité, qui n'était qu'un simple dispositif d'équité pour les salariés dont l'espérance de vie est plus courte et dont les conditions de retraite sont moins bonnes que celles des autres, que les nôtres, recul pour les salariés, et un gain, en revanche, non pas pour les petits patrons qui se préoccupent de leurs salariés, mais pour les grandes entreprises et leurs dirigeants. Mes chers collègues, ce texte manque vraiment d'équilibre. Pourquoi finalement ne pas l'appeler « projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances des mesures déstructurant le dialogue social » ? La parole

Je vous rappelle, chers collègues de gauche comme de droite, qu'il a été inscrit dans la loi sur les retraites de 2013 comme une contrepartie d'un nouveau recul de l'âge du départ à la retraite. Ce n'est donc pas un progrès social, mais un moindre mal, le salarié cumulant le maximum de points pouvant au mieux ne pas être pénalisé par la contre-réforme de 2013.

compte de certains facteurs de pénibilité, mais-c'était son atout principal -il devait favoriser la prévention plutôt que la réparation.

que 48 % des ouvriers sont exposés à un facteur de pénibilité et qu'un salarié sur huit, selon l'Agence nationale de santé publique, est exposé à un facteur cancérigène. Enfin, le nouveau dispositif sera financé dans le cadre de la branche AT-MP-

Le Gouvernement invoque la difficulté, pour les chefs de petites et moyennes entreprises, à faire face à ces nouvelles obligations, qui ne sont pas exemptes, il est vrai, d'une certaine lourdeur administrative. Qu'il faille entendre les difficultés de ces chefs d'entreprise, c'est une évidence. Mais, plutôt que d'imaginer un accompagnement par la puissance publique, le Gouvernement nous demande de l'autoriser à simplifier le compte pénibilité, mis en place sous le quinquennat précédent.

entendait le supprimer, car il « induit que le travail est une douleur », ajoutant que « le mot " pénibilité " ne correspond pas à ce dont nous avons besoin, parce que le travail c'est l'émancipation, c'est ce qui vous donne une place dans la société ». Le 8 juillet, en parfait accord avec cette déclaration, le Premier ministre a précisé la volonté présidentielle : le compte personnel de prévention de la pénibilité, bienvenue au compte professionnel de prévention. On sait l'attachement du Président de la République aux symboles, mais, en l'occurrence, le changement n'est pas que sémantique ... Ainsi, quatre des dix critères de pénibilité, ceux qui déplaisaient le plus au patronat,

Les salariés exposés à ces risques-là pourront encore bénéficier d'un départ anticipé à la retraite seulement quand « une maladie professionnelle a été reconnue » et quand « le taux d'incapacité permanente excède 10 % », précise la lettre du Premier ministre. En ces termes, comment accorder confiance au Gouvernement ? Par cette ordonnance, il entend donner pleine et entière satisfaction au MEDEF, sans considération pour la souffrance des 800 000 salariés déclarés au Je rappellerai au Président de la République, qui est féru de philosophie, que le mot « travail » vient du latin, qui désignait un instrument romain de torture destiné à punir les esclaves rebelles

Je souhaite m'arrêter sur la question de l'exposition aux risques chimiques, dont la déclaration et la mesure dans le compte pénibilité furent un progrès important du dernier quinquennat. « Cette avancée devait notamment contribuer à la prévention de ces maladies contractées au travail, qui, nous devons le rappeler, tuent encore régulièrement et ne font que rarement et dans une faible mesure l'objet de reconnaissance en tant que maladies professionnelles. « Le Premier ministre a indiqué aux organisations syndicales le sens de la réforme voulue les travailleurs soumis acquerront des " droits à départ anticipé à la retraite " s'ils développent une " maladie professionnelle " ayant été " reconnue " et entraînant un taux d'incapacité permanente supérieur à 10 %.

pouvoir bénéficier du dispositif ... « S'agissant des cancers professionnels, et plus généralement des " risques invisibles ", dont la matérialité n'est établie que lorsque s'en manifestent les effets, le problème essentiel réside dans le temps de latence entre l'exposition et l'apparition de la pathologie, laquelle survient souvent après la retraite le dispositif risque donc d'être peu opérant et extrêmement injuste. « Il risque en outre d'entretenir la faible connaissance des effets sanitaires et environnementaux de l'extrême contamination chimique dans l'activité au travail, laquelle contribue essentiellement à l'insuffisante protection des travailleurs et citoyens contre les risques chimiques. Le suivi lacunaire de l'exposition rend régulièrement impossible la détermination des causalités et des responsabilités dans l'empoisonnement. La très récente demande de non-lieu formulée par le parquet dans le volet pénal du dossier de l'amiante, en raison de la présumée

risques connus. « Plutôt que de poursuivre l'objectif de faire cesser le scandale de l'empoisonnement, parfois mortel, des travailleurs exposés à des agents chimiques sur leur lieu de travail,

il avait le grand mérite de reconnaître la pénibilité de certains travaux et de certains secteurs d'activité et ouvrait ainsi la voie à la responsabilité sociale de l'entreprise. Surtout, il visait à permettre aux salariés d'arriver à la retraite en bonne santé.

à la bonne performance de l'entreprise. Ainsi, le projet de loi prévoit d'autoriser le départ à la retraite anticipée des seuls salariés qui auront développé une maladie professionnelle et pour lesquels un taux d'invalidité de 10 % au moins aura été reconnu.

tout comme le transfert du financement à la branche AT-MP, qui n'a d'autre motif et n'aura d'autre effet que de déresponsabiliser les employeurs et d'alléger leurs obligations en matière de prévention, plus encore avec la réduction des moyens du CHSCT ou sa dilution dans la délégation unique du personnel, car l'on ne peut pas croire que cela se fera à moyens constants. Nous sommes loin du plan « santé au travail », qui tend à agir contre les risques professionnels prioritaires et à favoriser la prévention, en tant que levier de la performance des entreprises. Il s'agit d'un retour en arrière inquiétant pour la santé des travailleurs, substituant une logique de réparation à la logique de prévention. Pourtant, lorsqu'on voit les efforts du patronat pour s'exonérer de toute obligation en matière de protection des salariés,

Riocreux, sur l'article. Madame la ministre, je me fais le relais de notre collègue Anne Émery-Dumas, qui a dû nous quitter et qui souhaitait intervenir sur l'article 5, plus particulièrement sur l'alinéa 3 Comme l'indique à juste titre l'étude d'impact, en matière de détachement des travailleurs, le contexte est celui d'une augmentation constante du nombre de déclarations de prestations de services réalisées par des entreprises étrangères et des travailleurs détachés.

au niveau de l'inspection du travail, a permis l'augmentation sensible du nombre des déclarations. C'est donc un dispositif qui fonctionne bien et donne des résultats en matière de lutte contre le travail illégal et la fraude au détachement.

critères de pénibilité. Les salariés exposés au travail pénible doivent bénéficier de garanties, notamment en matière de départ à la retraite anticipée. Toutefois, il faut que les entreprises puissent appliquer les règles de mesure de la pénibilité ; or certaines d'entre elles sont totalement inapplicables par les TPE-PME.

par « des expositions aux agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques, des expositions à des facteurs de pénibilité- contraintes physiques marquées, environnement agressif, rythmes de travail contraints -et expositions à des facteurs de risque psychosociaux ». Selon ce même rapport, en 2010, plus de 8 millions de salariés français, soit près de 40 % du total, étaient exposés à au moins un facteur de pénibilité,

au moins économique à miser sur la prévention et à prendre soin des salariés. Le problème, c'est que cette logique, ou ce bon sens, n'est pas partagée par tous les chefs d'entreprise.

Je vous remercie, madame la ministre, pour les éclaircissements complémentaires apportés aujourd'hui. La pénibilité est un véritable sujet. Devoir subir une succession de prises de parole répétitives sur l'article 5 en a été une illustration pour certains d'entre nous Personne ne remet en cause la difficulté de certains métiers et ses conséquences potentielles sur la santé. Mais plutôt que d'essayer à tout prix de déterminer le degré de pénibilité salarié par salarié, tâche par tâche, il faut améliorer les conditions de travail et la prévention. C'est le choix de l'Allemagne et des pays scandinaves, notamment. En cas de métier pénible, devenu dangereux l'âge avançant, il faut privilégier le reclassement dans un emploi moins rude, toujours grâce à la formation. La France fait le choix de prévoir des départs anticipés à la retraite. On attend le dernier moment pour agir, en indemnisant plutôt qu'en protégeant. La pénibilité d'une carrière pourra évidemment être prise en compte pour un départ anticipé à la retraite, mais cela impliquera, pour assurer la pérennité du système, que les régimes spéciaux soient entièrement revus, car il n'est plus acceptable que des salariés bénéficient de conditions de départ en retraite plus que favorables sans avoir exercé un métier plus pénible qu'un autre, quand d'autres doivent attendre plusieurs années supplémentaires pour accéder à une retraite à taux plein.

Le code du travail précise que « le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

2000-2012 indiquait que le nombre de contrats à durée déterminée avait progressé de plus de 75 % en France. En dix ans, le nombre de CDD de moins d'un mois de CDD de moins d'un mois a plus que doublé, passant de 1,8 million à 3,7 millions entre les troisièmes trimestres de 2003 et de 2013. Certes, le CDI reste le contrat de travail le plus représentatif du salariat en France, mais une majorité des embauches se font donc désormais en CDD. Ces contrats temporaires touchent surtout les jeunes et les moins qualifiés, avec toute la précarité que cela entraîne. Compte tenu de ces éléments, et puisque vous avez l'ambition de modifier le code du travail pour apporter plus de protection aux salariés, nous vous proposons d'adopter notre amendement, qui vise à limiter le recours aux CDD à des cas précis. Nous souhaitons qu'ils cessent d'être utilisés comme des variables d'ajustement des entreprises, qui dérogent allègrement à la réglementation en les substituant très souvent à des emplois permanents.

la mise en place de critères collectifs de reconnaissance de la pénibilité dans chaque branche, remplaçant les fiches individuelles qui rendent complexe la prise en compte de la pénibilité et permettant, en fonction du nombre de critères de pénibilité dans chaque métier- travail de nuit, horaires décalés, chaleur, vibrations ...

et dont Mme la ministre vient de préciser les modalités. Nous considérons que cette réforme est indispensable, mais elle ne doit pas pour autant conduire à remettre en cause le principe d'une prévention et d'une compensation de la pénibilité.

L'alinéa 3 porte surtout sur l'adaptation de la législation du travail détaché à certaines spécificités. On ne peut néanmoins voter ce projet de loi d'habilitation sans traiter du sujet d'ensemble. Alors que l'Europe travaille en ce moment même à une refonte de sa directive sur le travail détaché, nous n'avons de fait aucune garantie que les demandes portées par la France seront satisfaites, qu'il s'agisse du contrôle à la source de l'entreprise qui envoie des travailleurs détachés, de la réduction de la durée du détachement, détachement, du cabotage ou des sociétés boîtes aux lettres. Madame la ministre, c'est le principe même de la directive européenne sur le travail détaché qui doit être revu. Il n'est pas acceptable que des entreprises qui envoient des salariés détachés en France ne paient pas les cotisations sociales qui sont exigées des entreprises françaises.

de préciser quelque peu ses orientations en la matière. Cette habilitation est destinée à faciliter les démarches administratives pour les travailleurs détachés frontaliers. Les craintes que vous aviez, mon cher collègue, auront certainement été apaisées par par les propos de Mme la ministre. Je vous invite donc à retirer cet amendement, faute de quoi la commission sera obligée d'émettre un avis défavorable. Pour ce qui est de l'amendement n° 233, le Gouvernement souhaite élargir le champ d'habilitation relatif aux travailleurs frontaliers. Il désire en effet assouplir les règles de détachement applicables aux entreprises étrangères qui réalisent régulièrement de courtes prestations sur le territoire national. Sont notamment visés les sportifs, encore les scientifiques. Le renforcement des règles relatives à la déclaration préalable de détachement issu de la loi dite « Savary » du 10 juillet 2014 permet d'améliorer la lutte contre les fraudes

ou alternativement, sur la subordination juridique et la dépendance économique. Notre amendement vise aussi à encadrer le recours à la sous-traitance par sa limitation légale à deux degrés et son contrôle par les travailleurs. Le recours à la sous-traitance serait soumis à l'avis conforme du comité d'entreprise, qui a toute compétence pour apprécier les besoins et possibilités de l'entreprise.

La loi El Khomri a profondément réduit les capacités de la médecine du travail. Au motif du manque de praticiens, le gouvernement dirigé par Manuel Valls avait décidé de réduire des visites médicales jugées trop nombreuses et trop souvent inutiles, plutôt que de s'attaquer aux raisons de la pénurie de médecins du travail. Notre amendement vise à revenir sur cette modification de la médecine du travail, qui prévoit un suivi attentif uniquement pour les salariés exerçant des métiers dits « pénibles ». Nous ne pouvons que nous étonner d'une telle conception de la médecine du travail, qui ne serait plus là pour veiller à la santé de tous les travailleurs. Permettez-moi de revenir

le médecin du travail devrait être, avec le CHSCT, le plus à même de constater les troubles physiques et psychiques des salariés. Combien faudra-t-il de drames ? Je pense notamment

59. L'article 6 habilite le Gouvernement à modifier le code du travail en vue d'harmoniser l'état du droit pendant douze mois après la promulgation du présent projet de loi. Sous couvert de coordination et de mise en cohérence rédactionnelles, cet article laisse de trop grandes marges de manoeuvre, selon nous, au Gouvernement pour modifier le code du travail sur le fond, les réécritures du code étant rarement faites à droit constant. Pour ces raisons, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article. Merci L'article 6 habilite le Gouvernement à modifier le code du travail en vue d'harmoniser l'état du droit pendant douze mois après la promulgation du présent projet de loi. Cette habilitation très large laisse au Gouvernement une marge de manoeuvre excessive, des modifications notables du code du travail pouvant être introduites au nom de la mise en cohérence des textes. Compte tenu de l'objet du texte, qui touche aux bases mêmes du droit social, une habilitation aussi vague dessaisit à l'excès le Parlement. Pour ces raisons, je propose la suppression de cet article. présenter l'amendement n° 85 rectifié . Cet article autorise le Gouvernement à harmoniser l'état du droit, à assurer la cohérence des textes, à abroger les dispositions devenues sans objet et à remédier aux éventuelles erreurs.

cet article laisse de grandes marges de manoeuvre au Gouvernement pour modifier le code du travail sur le fond, les réécritures du code étant rarement faites à droit constant. Pour

? Je comprends bien l'intention des auteurs de cet amendement, mais l'habilitation prévue à l'article 6 ne permet pas au Gouvernement de modifier le fond du droit.

les moyens d'assurer la bonne insertion dans notre ordre juridique des modifications apportées par les ordonnances, ne peuvent mécaniquement pas se faire à droit constant par rapport à la situation actuelle, c'est-à-dire antérieure à la publication des ordonnances. Par conséquent, la commission demande le retrait

Cohen, sur l'article. L'article 7, tel que modifié par la majorité sénatoriale en commission, prolonge la période transitoire relative à la mise en place du nouveau zonage dérogatoire

Les sociologues Laurent Lesnard et Jean-Yves Boulin ont publié une enquête très intéressante intitulée « Travail dominical, usages du temps et vie sociale et familiale », », qui analyse les conséquences du travail dominical sur la vie personnelle des salariés du privé et des fonctionnaires mobilisés ce jour-là. Hors agriculture, on estimait à 6,5 % la part de la population active qui travaillait le dimanche en 1970. En 2010, cette proportion est passée à 14 %. Elle ne cesse d'augmenter. Nous sommes face à un renversement que l'on peut qualifier d'historique

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Au regard de l'application d'ordonnances remettant en cause les modalités de négociation des accords et conventions dans le domaine salarial, il convient que cette prorogation

Le parallélisme des formes doit être rétabli. Dès lors que des organisations syndicales représentatives peuvent demander au préfet l'abrogation de l'arrêté, il est logique de prévoir que les organisations syndicales demandant au préfet l'adoption de cet arrêté soient, elles aussi, représentatives.

sujet technique. Cet amendement vise à ajouter une condition à l'édiction des arrêtés préfectoraux de fermeture dominicale prévue à l'article L. 3132-29 du code du travail. Les accords sur lesquels ils s'appuient devraient être conclus par des organisations représentatives. Une telle mesure est difficilement applicable, car les périmètres des arrêtés de fermeture sont aujourd'hui départementaux et infradépartementaux. La profession

des dernières lois majeures relatives au droit du travail. Dans la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, le Gouvernement s'était engagé à remettre au Parlement quinze rapports, le dernier au plus tard le 31 décembre 2015. Seuls deux nous ont été communiqués. Aucun des cinq rapports prévus par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale n'a été transmis au Parlement. pour les trois rapports prévus par la loi Rebsamen du 17 août 2015. Enfin, ce sont déjà cinq rapports prévus par la loi El Khomri du 8 août 2016 qui sont en retard. Je vous informe d'ailleurs, madame la ministre, que vous devez transmettre au Parlement, avant le 8 août prochain, un rapport dressant le bilan de la mise en oeuvre de la base de données économiques et sociales- c'est l'article 20 de la loi El Khomri -, un rapport sur l'état des discriminations syndicales en France- c'est l'article 30 -, ainsi qu'un rapport présentant des propositions pour renforcer l'attractivité de la carrière de médecin du travail- c'est l'article 104. Je peux dire, à titre d'exemple, que nous espérons toujours obtenir un jour le rapport sur l'articulation entre le code du travail et les statuts des personnels des chambres consulaires, qui aurait dû être remis le 31 décembre 2013, en application de l'article 26 de la loi du 14 juin 2013, ou encore celui sur la redéfinition, l'utilisation et l'harmonisation des notions de jour dans le code du travail, que je sais cher à Nicole Bricq et qui aurait dû nous être remis avant le 9 mai dernier en application de l'article 13 de la loi El Khomri. Je tiens enfin à lever un malentendu qui est apparu

fait mention d'un rapport, très utile d'ailleurs, sur ce thème. Il s'agit toutefois non d'un rapport du Gouvernement au Parlement, mais du résultat de la concertation engagée par les partenaires sociaux en application de l'article 57 de la loi El Khomri. C'est l'occasion de souligner, pour conclure, que ce même article prévoyait que le Gouvernement remettrait au Parlement avant le 1 décembre 2016 un rapport sur l'adaptation juridique des notions de lieu,

31 décembre 2017, d'un rapport d'évaluation des dispositifs de sécurisation de l'emploi existants et des axes d'amélioration, en vue de mettre en place une sécurité sociale professionnelle pour tous les salariés.

2017, cet amendement vise à lancer le débat sur la mise en oeuvre d'une véritable sécurité sociale professionnelle pour tous.

lorsqu'il se prolonge que pour des raisons psychologiques et sociétales. Il induit un sentiment d'humiliation, la perte d'estime de soi, la peur du regard des autres, la perte des savoir-faire. Le nombre de suicides liés au chômage est considérable. Selon

éducative- quand on a perdu l'estime de soi, on ne peut plus s'intéresser aux autres, en particulier à ses enfants -, et peuvent entraîner des conduites addictives et l'exclusion sociale. Le maintien d'un lien avec l'entreprise, lorsque celle-ci n'a pas disparu, permettrait

qui leur permet justement de rester liés contractuellement à leur entreprise d'origine pendant leur formation. Toutefois, une telle obligation ne pourrait pas être généralisée à toutes les entreprises en deçà de ce seuil. Je crois savoir que le Gouvernement et les partenaires sociaux souhaitent améliorer le contrat de sécurisation professionnelle auquel ont droit tous les salariés licenciés pour motif économique dans les entreprises de moins de 1 000 salariés. Peut-être souhaiteront-ils explorer la piste ouverte par M.

d'autre solution que de vous demander un rapport sur la situation, au regard de l'assurance chômage, des agents non titulaires français recrutés localement par les administrations françaises à l'étranger. Ces personnels représentent, par exemple, environ un tiers des 4 500 recrutés locaux du ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Leur nombre va croissant à mesure que les postes d'expatrié sont supprimés. À leur retour en France, les recrutés locaux-contrairement aux agents détachés à l'étranger ou expatriés -se voient refuser le bénéfice d'une allocation d'assurance chômage, qu'il s'agisse de l'allocation temporaire d'attente, l'ATA, ou de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, Or, en vertu de l'article L. 5424-1 du code du travail, l'État et ses établissements publics administratifs ont l'obligation d'assurer leurs agents non fonctionnaires contre le risque de privation d'emploi. Dans une décision du 27 février 2013, le Défenseur des droits considère que les recrutés locaux « subissent une différence de traitement qui n'apparaît pas justifiée tant au regard de la situation des agents non titulaires de l'État, que de celle des salariés du secteur privé placés dans une situation comparable Il recommande donc au Gouvernement de « prendre les mesures nécessaires en vue de permettre à ces agents [ ...] de bénéficier des droits à indemnisation chômage à leur retour sur le territoire français ». Force est malheureusement de constater qu'aucune suite positive n'a encore été donnée à cette recommandation, qui va dans le même sens qu'un télégramme diplomatique en date du 9 septembre 2009, selon lequel l'ouverture des droits à l'assurance chômage « s'applique [ ...] aux ADL- agents de droit local -qui décideraient de venir résider en France dans les douze mois qui suivent la fin de leur contrat En déposant cet amendement, nous souhaitons que le Gouvernement indique au Parlement comment il entend améliorer le régime de protection sociale des personnels de droit local, qui jouent un rôle central dans le fonctionnement des postes diplomatiques et consulaires, des instituts culturels et des établissements scolaires français. Toutes les pistes doivent être explorées, y compris l'auto-assurance, la conclusion d'une convention de gestion avec Pôle emploi et l'adhésion individuelle au régime français d'assurance chômage. Madame la ministre,

J'espère que la ministre pourra y apporter une réponse. Je lui en souffle une : je pense que si nous adoptions cet amendement, aucun rapport ne verrait jamais le jour

le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi pour sécuriser la situation des agents non titulaires de droit local et leur permettre de bénéficier d'une indemnisation au titre de l'assurance chômage.

Entre certaines situations aujourd'hui insupportables, indignes pour les salariés ou défavorables au développement économique et le monde idéal dont nous avons tous une vision et dont nous rêvons, il existe- c'est ma conception de l'action politique -un champ

Parmi les nombreux reculs que comporte le texte, nous citerons le plafonnement des indemnités de licenciement, la suppression du compte pénibilité, la réduction des délais de recours aux prud'hommes, la fusion des instances représentatives du personnel. Non, mes chers collègues, il n'est pas difficile de licencier en France ! Non, les contraintes qui pèsent sur les entreprises ne sont pas trop rigides, notamment en matière de licenciement.

qu'on ne peut tout de même pas soupçonner de complaisance à l'égard de notre modèle social, rappelle même qu'il est plus facile de faire un plan social en France qu'en Irlande, en Hongrie, en Allemagne, en Suisse, en Italie, en Belgique, parmi d'autres pays. Malgré ces éléments objectifs,

d'étendre à de nombreux domaines l'inversion de la hiérarchie des normes et la suppression du principe de faveur, avec toutes les inégalités que cela va engendrer, de rendre la loi supplétive, voire accessoire, de généraliser la précarité en créant des CDI

La raison en est simple : le travail structure nos vies et celles de nos concitoyens. Deux visions s'opposent sur le droit du travail : d'aucuns le souhaitent centralisé, légal, exhaustif ; d'autres, dont je fais partie, veulent faire confiance à l'intelligence collective.

Madame la ministre, c'est maintenant à vous de jouer. La partie sera difficile. Soyez ferme face à ceux qui cherchent à vous déstabiliser. Ne reculez pas devant les dogmatismes et les vieilles lunes. Il y aura de nombreuses résistances, peut-être violentes, comme nous avons pu en voir l'an dernier. Accrochez-vous aux principes qui doivent guider votre réforme. Placez le dialogue social au plus près de l'entreprise, au plus près du terrain. Fluidifiez le dialogue social dans les entreprises, un dialogue direct, sans intermédiaires obligatoires. Simplifiez les règles applicables aux administrations et adaptez le rôle de celles-ci. Enfin, flexibilisez le marché du travail pour permettre aux entreprises de s'adapter. Nous nous reverrons prochainement pour parler de formation professionnelle, d'assurance chômage, de retraites.

Vite, vite, vite : vous le devez, nous le devons aux entreprises, à celles et à ceux qui contribuent à leur réussite, ainsi qu'aux chômeurs qui souhaitent retrouver un emploi. Bon courage

Vous ne pouvez pas l'instaurer à tous les étages de la démocratie sociale si vous n'acceptez pas le principe de l'accord majoritaire.

que les règles habituelles de la démocratie parlementaire ne soient pas respectées. Au Sénat, nous les respectons

la courbe du chômage. Madame la ministre, mes derniers mots seront pour vous : j'ose espérer que, à l'inverse de vos prédécesseurs, vous aurez trouvé les bonnes réponses ; pour les salariés, j'espère que vous avez raison.